Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, permettant une bonne application du régime d'asile européen. Je rappelle que la discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte

suivront, marquer notre profond désaccord tant avec l'esprit qu'avec la lettre de cette proposition de loi. Permettez-moi de faire une première remarque sur le. Examinée, et probablement adoptée, à quelques semaines des débats sur le projet de loi

Priver de liberté des personnes en situation régulière sur le territoire français est, mes chers collègues, contraire à nos principes fondateurs et viole, sans nul doute, l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme. Comme l'observe Amnesty International, dont nous partageons les préoccupations, le texte cherche à « sauver » le règlement Dublin en le renforçant, alors que ce dernier se révèle depuis des années vain, inéquitable et inefficace. De surcroît, la proposition De surcroît, la proposition de loi porte gravement atteinte au droit d'asile lui-même et au respect des obligations internationales de la France à cet égard. Elle vise en effet à placer en rétention des personnes dont les empreintes apparaîtraient dans le fichier EURODAC avant même qu'elles n'aient pu enregistrer leur demande d'asile, bafouant ainsi un droit fondamental. Peut-on, sans sourciller, voter un texte d'une telle nature ? Nous ne le pensons pas, bien entendu. Nous ne sommes d'ailleurs pas totalement isolés puisque, en dehors des ONG internationalement reconnues et des très nombreuses associations qui dénoncent les dérives de ce texte, le Défenseur des droits lui-même n'a pas eu de mots assez forts pour dire sa préoccupation à l'égard de cette proposition

et enregistre la plupart des personnes qui entrent sur le territoire de l'Union européenne. Si nous voulons être du côté de ceux qui veulent une politique de l'asile solidaire

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande Le scrutin est ouvert.

Or aucune définition de la vulnérabilité ne figure dans l'article, ce qui laisse une grande marge d'appréciation à l'administration. Dans le cas précis de la procédure que nous examinons aujourd'hui, laquelle vise à placer en rétention administrative des personnes demandant l'asile à partir d'un simple faisceau d'indices,

Le texte vise précisément « les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines Il me semble que ces critères sont sensiblement les mêmes que ceux qui devraient s'imposer aux services administratifs au moment de la décision de placement. C'est pourquoi il m'a semblé raisonnable de faire référence à l'article susmentionné. Je souhaiterais que l'on m'indique où figure la définition de la vulnérabilité des personnes concernées par le placement en rétention avant qu'une décision de transfert ne soit prise contre elles.

L'objet de cet amendement est simplement de faire en sorte que ne soient pas placés en rétention administrative des demandeurs d'asile sans que ceux-ci aient la certitude qu'ils feront l'objet d'une procédure de transfert, ce qui est une nouveauté introduite par la En effet, le texte proposé par nos collègues de l'Assemblée nationale comporte le risque de placer en rétention des personnes éligibles à une protection internationale. Sommes-nous prêts à prendre ce risque ? ce risque ? Il me semble que nous devrions d'abord être en mesure de l'évaluer. Or tel n'est pas le cas aujourd'hui. Notre rapporteur a reconnu, d'une part, qu'il était difficile d'élaborer des statistiques nationales consolidées pour fixer une estimation raisonnable du nombre de « dublinés » susceptibles d'être ainsi mis en rétention, critère par critère, et, d'autre part, que les capacités d'accueil actuelles des centres de rétention administrative ne suffiraient pas. le placement en rétention administrative et les procédures de transfert sous escorte ont un coût foncier et d'encadrement non négligeable, si l'administration choisit de placer en rétention des demandeurs d'asile dès leur demande, et ce jusqu'à la réalisation du transfert. Dans les cas où l'État responsable se montre peu coopératif, ce qui reste trop fréquent selon le rapport, les durées de rétention pourraient être très longues. Je ne sous-estime pas les difficultés auxquelles font face les forces de l'ordre, mais je crains qu'une possibilité de rétention encore plus précoce ne conduise ces personnes à choisir un peu plus la clandestinité. Là encore, il ne s'agit pas d'entêtement : j'attends d'être convaincue plutôt que persuadée ... Sur un sujet aussi grave, nous ne devrions pas nous contenter de conduire une politique au doigt mouillé. Quel est

défavorable. Cet amendement tend à limiter le placement en rétention à l'étranger ou au demandeur d'asile qui s'est vu notifier une décision de transfert et de l'interdire pendant la phase de détermination de l'État responsable. Sur ce point, la proposition de loi ne fait que mettre en oeuvre les dispositions de l'article 28 du règlement Dublin. En effet, pour garantir l'efficacité des transferts, le droit européen permet de placer en rétention l'ensemble des étrangers faisant l'objet d'une procédure Dublin, quelle que soit l'étape de la procédure. Notre législation nécessitait d'être précisée quant aux modalités de mise en oeuvre de ces dispositions

est ainsi libellé : La parole est à Mme Josiane Costes. Cet amendement vise à prendre en considération les voies de recours qui existent devant les juridictions de l'État responsable dans l'évaluation du risque de fuite d'un demandeur d'asile en vue d'une procédure de transfert. En France, par exemple, près de 17 % des décisions de refus d'octroi d'une protection de l'OFPRA ont été annulées par la Cour nationale du droit d'asile en 2017. On peut considérer que le risque non négligeable de fuite est établi dès lors que le demandeur d'asile perd l'espoir d'une acceptation de sa demande. Tel n'est pas le cas des personnes ayant introduit un recours contre une décision de refus. Cet amendement vise également à protéger l'autorité de la chose jugée des décisions juridictionnelles de nos partenaires européens, une notion importante dans un État de droit, à laquelle beaucoup d'entre nous sont attachés. tend aussi à ne pas exposer des personnes qui se verront accorder l'asile à des mesures de rétention administrative, et de limiter celles-ci aux cas les plus évidents, conformément à l'esprit de l'article 28 du règlement Dublin III. Quel est l'avis de la commission ?

donc défavorable. Je signale à la Haute Assemblée que l'adoption de cet amendement interdirait le placement en rétention en France d'un migrant sous statut Dublin débouté du droit d'asile, mais n'ayant pas épuisé les voies de recours devant la juridiction de l'État membre responsable de l'analyse.

doit y rester même si sa demande d'asile est rejetée en première instance. D'ailleurs, s'il se rend dans un autre pays, par exemple en France, après avoir été débouté en Allemagne, il se sait dans l'illégalité et pourrait donc être tenté de fuir le territoire national. Enfin, la proposition de loi

également défavorable. En effet, l'épuisement des voies de recours n'a aucun lien avec la définition du risque non négligeable de fuite. Ce critère ne figure pas au nombre de ceux qui sont exigés par les règlements Dublin pour déterminer l'État membre du traitement de la demande d'asile. En outre, les voies et délais de recours contre la décision de refus d'octroi d'une protection internationale relèvent des dispositions de la directive Procédure et sont sans effet sur l'application du règlement Dublin. La parole

La liste des critères initialement retenus pour établir le risque non négligeable de fuite a été étoffée lors de l'examen de la proposition de loi par l'Assemblée nationale. Parmi les critères prévus figure le fait pour le demandeur d'asile de s'être soustrait à des mesures d'éloignement de droit commun. Le rapport de M. Buffet montre que l'application de la procédure de transfert permise par le règlement Dublin est progressivement montée en puissance pour concerner 15 %, puis 30 % des demandeurs d'asile sur notre sol. Par souci d'efficience administrative plus que d'efficacité, nous considérons que, dans l'intérêt des demandeurs d'asile, des forces de l'ordre chargées d'appliquer ces mesures et, une fois encore, des contribuables, l'autorité administrative devrait s'astreindre à ne pas multiplier les fondements d'expulsion d'un demandeur d'asile et s'employer

Nous craignons que la reconnaissance de la non-soumission à une autre mesure d'éloignement comme indice de l'existence d'un risque non négligeable de fuite en vue de la mise en oeuvre d'une procédure de transfert ne conduise, dans le premier cas, à disperser inefficacement l'action du Gouvernement. Pour paraphraser Montesquieu, prenons garde que les actes administratifs inutiles n'affaiblissent les actes administratifs nécessaires ... Quel est l'avis de la commission ?

évidemment défavorables, car une même personne peut se voir imposer une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, s'y soustraire puis déposer une demande d'asile, alors qu'un autre État est responsable de l'examen de cette demande. La loi doit évidemment prévoir de tels cas de figure. Nous savons tous combien l'imagination peut être grande ... Enfin, la notion de mesure d'éloignement doit être conservée : elle est suffisamment large pour englober à la fois les OQTF et les mesures d'ordre public, comme les interdictions de circulation sur le territoire national et les expulsions pour motif d'ordre public. Quel est l'avis du Gouvernement ?

au moins équivalent à la lutte contre le vagabondage d'étrangers sur notre sol. Pourtant, cette réalité des migrations contemporaines est largement sous-estimée dans le traitement actuel des demandes d'asile et de l'immigration illégale, comme nous l'avons récemment souligné dans le débat sur les mineurs non accompagnés. Le règlement Dublin III est d'ailleurs muet sur ce point, à l'exception de son article 6, consacré aux garanties en faveur des mineurs. L'article L. 744-6 du CESEDA, consacré à l'évaluation de la vulnérabilité par les agents de l'OFPRA, que j'ai cité précédemment, fait expressément référence à la traite des êtres humains. Cet amendement a pour objectif de contraindre l'administration, dans ses démarches en présence de demandeurs d'asile, à mieux prendre en compte cette réalité, dès le premier stade de la procédure. En effet, l'existence de réseaux de passeurs contribue incontestablement à accroître la mobilité des demandeurs d'asile dans l'Union européenne, les premiers distillant des informations erronées susceptibles de causer préjudice aux seconds. Ces réseaux encouragent également les demandeurs d'asile comme les migrants économiques à franchir les frontières illégalement plutôt qu'à recourir aux dispositifs légaux existants, tels que les visas humanitaires. La lutte contre la traite des êtres humains par des réseaux de passeurs devrait donc devenir une priorité en France et dans l'Union européenne ! Quel est l'avis de la commission ?

4 et 21. De plus, le texte prévoit déjà expressément que l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité ne pourra constituer, à elle seule,

? Je précise à Mme Costes que le Gouvernement lutte avec beaucoup de fermeté contre les réseaux de passeurs

contrairement à ce que prévoit le critère suivant, le critère g). Cet amendement vise à souligner l'absurdité d'une disposition qui aurait pour effet d'encourager la création de nouvelles places en centres de rétention administrative plutôt que des places d'hébergement normales. Je considère au contraire que l'augmentation des capacités des centres d'hébergement doit rester la priorité, ne serait-ce que pour pouvoir localiser au mieux les personnes ayant formulé une demande d'asile, ce qui n'est d'ailleurs pas contraire à la volonté du Gouvernement de recourir à des assignations à résidence en vue d'un transfert.

une personne est prise en charge à son entrée sur le territoire français commence par un hébergement. En sorte que les personnes dont nous parlons sont des personnes qui, après être entrées dans un hébergement offert

il peut s'agir pour eux d'échapper à l'exploitation de tels réseaux plutôt qu'à la décision de transfert vers l'État responsable de leur demande d'asile. L'amendement n° 13 rectifié,

précision. Quel est l'avis de la commission ?

population mineure en rétention : « Entre 2014 et 2015, le nombre des mineurs placés en rétention administrative avec leurs parents était passé de 45 à 105, ce qui représente une augmentation supérieure à 133 %. La situation est encore plus inquiétante dans les locaux de rétention administrative, les LRA. Comme le souligne l'article 3 de ce texte, les centres de rétention administrative sont des lieux où l'on croise des individus aux parcours très variés demandeurs d'asile, mais également étrangers expulsés à des fins d'ordre public. La police aux frontières, qui encadre les centres de rétention administrative, n'est pas spécifiquement formée à l'accueil de si jeunes publics et de familles. de privation de liberté dans son récent rapport consacré au personnel des lieux de privation de liberté : « Dans les centres de rétention administrative, l'administration comme les organisations professionnelles soulignent un décalage important entre les missions de police liées aux fonctions judiciaires ou de sécurité publique, principalement mises en avant au cours de la formation initiale, et les missions en centre de rétention administrative. De ce point de vue, le fait d'avoir à priver de liberté des personnes qui ne sont pas délinquantes, parfois même des enfants, est un poids psychologique que plusieurs interlocuteurs du CGLPL ont souligné. À cette difficulté de principe s'ajoute celle qui consiste à placer en environnement clos des fonctionnaires qui ont parfois choisi le métier de policier pour la liberté de mouvement qu'il confère. La fonction de surveillance elle-même peut alors être regardée comme aliénant la liberté de celui qui l'exerce. Le règlement Dublin III fait lui-même expressément référence à la convention internationale des droits de l'enfant et au respect de la vie familiale des demandeurs d'asile, aux paragraphes 13 et suivants. C'est pourquoi nous souhaitons que le placement en rétention des mineurs soit limité à un délai très court, explicitement prévu par la loi. Tel est l'objet de cet amendement.

et des mineurs qui les accompagnent. Or la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a fait de la rétention des personnes accompagnées de mineurs une mesure exceptionnelle, limitée à certains cas, notamment à celui des familles qui se sont soustraites systématiquement aux mesures d'éloignement.

En particulier, la durée du placement en rétention doit être la plus brève possible, sous le contrôle du juge. Fixer dans la loi un délai paraît donc peu opportun à ce stade.

au titre du 1° du I de l'article L. 561-2 que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable